depuis plusieurs années, la fiscalisation des majorations de pension et le gel des pensions. Nous demandons simplement la suppression de cette disposition qui va affecter le pouvoir d'achat des retraités, déjà pénalisés dans le présent projet de loi.

Présenté comme une mesure de simplification qui améliore la lisibilité du dispositif, ce décalage fait en réalité perdre une année de revalorisation aux retraités. Après l'augmentation de 1,7

sociale pour 2018 prévoit de reporter la date de revalorisation des pensions de retraite du 1 octobre au 1 janvier et d'avancer celle de l'allocation de solidarité aux personnes âgées du 1 avril au 1 janvier. Le décalage de trois mois des pensions de retraite fait perdre une année de revalorisation aux retraités. Cette mesure d'économie, qui vient s'ajouter à la hausse de la CSG, va renforcer la dégradation du pouvoir d'achat des retraités. Cet amendement vise donc à supprimer le report de trois mois de la date de revalorisation des pensions de retraite.

Dans une société en pleine mutation, la question des retraites ne peut pas être éternellement abordée sous le seul angle paramétrique. En 2010, lors de l'examen du projet de loi portant réforme des retraites, plusieurs groupes, dont le RDSE, avaient demandé qu'une réflexion nationale soit organisée sur le principe d'une réforme systémique des retraites. Cette proposition faisait écho à un rapport du Conseil d'orientation des retraites de la même année selon lequel le passage d'un régime en annuités à un régime en points ou en comptes notionnels était techniquement possible et nous permettait notamment d'intégrer des dispositifs de solidarité. Nous sommes convaincus qu'une réforme systémique de la prise en charge collective du risque vieillesse est inévitable. Une telle évolution ne remet bien évidemment pas en cause le système de retraite par répartition auquel les Français sont profondément attachés. Ainsi, notre amendement tend à fixer un calendrier pour la mise en oeuvre d'une réforme systémique

Monsieur le rapporteur, madame la ministre, nous vous entendons. Je veux simplement rappeler ici que 2010-2017, c'est un septennat. S'il

efficacité ne fait aucun doute, et si l'on doit mettre en balance le bénéfice et le risque, le plateau penche nettement en faveur du bénéfice.

-dont l'imputabilité n'est pas prouvée, et des millions de vaccins administrés dans le monde avec une couverture excellente, il n'y a pas photo

Chers collègues, cette obligation, que beaucoup critiquent et dénoncent comme une renonciation d'autonomie, comme une altération de la liberté, ne sera effectivement coercitive que pour la frange qui refuse d'effectuer un geste altruiste visant à protéger non seulement ses enfants, mais aussi ceux des autres. La

L'article 34 prévoit de rendre obligatoires onze vaccins à partir du 1 juin 2018, pour tous les enfants nés à compter du 1 janvier de la même année. Cette mesure s'inscrit dans un contexte de recrudescence de certaines maladies et de foyers épidémiques- notamment la rougeole -et fait suite au rapport de Sandrine Hurel sur la politique vaccinale, remis en janvier 2016, et à une consultation citoyenne lancée en janvier 2016 par l'ancienne ministre des affaires sociales et de la santé, Marisol Touraine. Le Gouvernement a tranché et rend obligatoires onze vaccins, sans clause d'exemption. Quelques remarques me paraissent nécessaires. les vaccins seront obligatoires pour toute admission ou maintien dans une école, colonie de vacances ou autre collectivité d'enfants. Je considère que l'éviction scolaire n'est pas une solution et constitue une sanction lourde de conséquences pour les enfants concernés qui se verront, par la force des choses, marginalisés et mis au ban de la société dès leur plus jeune âge. Ensuite, avec la suppression de l'article L. L. 3116-4 du code de la santé publique, ce serait l'article 227-17 du code pénal qui s'appliquerait. Je me doute que ce type de poursuites ne serait pas à exclure, et même au « cas par cas », cette situation me préoccupe.

myofasciite à macrophages, maladie d'Alzheimer, maladie de Parkinson, maladie de Crohn, sarcoïdose ... De plus, certaines autorités sanitaires françaises, tout comme la justice, reconnaissent peu à peu que l'aluminium utilisé comme adjuvant dans les vaccins peut engendrer des effets secondaires graves : le Conseil d'État a ainsi reconnu le lien entre myofasciite à macrophages et aluminium vaccinal à huit

Il s'agit donc d'étendre la protection de l'ensemble des enfants de France contre des maladies fréquentes et potentiellement graves- méningite à pneumocoque ou méningocoque, rougeole, rubéole, coqueluche, hépatite B -pour lesquelles la couverture vaccinale reste très insuffisante. Je voudrais rappeler que 10 nouveau-nés sont morts de la coqueluche en 2015, 50 enfants et adultes d'une infection à méningocoque et plus de 1 000 adultes d'une hépatite.

Je le rappelle, l'aluminium est présent dans le chocolat, les tisanes et les déodorants. La vaccination a une double vocation de santé publique et de protection individuelle. L'obligation d'effectuer trois vaccins

En vous appuyant sur la concertation citoyenne présidée par le professeur Fischer, dont plusieurs participants ont dénoncé le caractère orienté et partial des conclusions, vous avez choisi le passage en force sur un sujet extrêmement sensible. Notre pays est le pays de Pasteur, le pays des vaccins, des vaccins, avancée scientifique majeure, qui a permis et permet encore d'éviter des morts, des contagions, des maladies graves. Je ne suis pas de celles et de ceux qui prônent une liberté vaccinale. Je suis résolument en faveur de la vaccination, mais cela fait des années que je m'interroge sur le contenu de certains vaccins. J'ai déjà eu l'occasion de le dire dans cet hémicycle, sans que cela trouve de résonance auprès du gouvernement de ce quinquennat ou du précédent, il est urgent d'informer objectivement nos concitoyens, notamment sur la présence et la nocivité de sels aluminiques utilisés comme adjuvants.

Vous remettez en cause le caractère nocif des sels aluminiques comme adjuvant. J'ai assisté, comme d'autres, à énormément de conférences sur le sujet. Pour ma part, madame la ministre, puisqu'il y a cette émotion, puisque des travaux sérieux, pas seulement français, ont été faits

C'est une recommandation de l'Organisation mondiale de la santé, qui en fait un objectif principal de son action dans les années qui viennent : il s'agit d'assurer une couverture vaccinale de 95 % de la population mondiale, de façon à éviter que des milliers d'enfants meurent ou restent handicapés.

avec le temps, dans les vaccins et qu'il n'était plus nécessaire de les rendre obligatoires. Ainsi, la plupart des parents pensent que les vaccins recommandés sont facultatifs, alors qu'ils sont totalement nécessaires à la protection de nos enfants, ceux qui peuvent être vaccinés et ceux qui ne peuvent pas l'être.

et indispensables à la santé des enfants. Enfin, je terminerai en disant qu'il s'agit d'un intérêt individuel pour tous les enfants qui sont vaccinés, mais également d'un intérêt collectif pour tous ceux qui sont malades et ne peuvent pas être vaccinés. Je pense notamment aux enfants atteints de cancer, qui, du fait d'un déficit immunitaire,

je voudrais au contraire souligner que cette concertation, qui a été longue, s'est déroulée en plusieurs phases avec, d'un côté, un panel de citoyens et, de l'autre côté, des professionnels de santé. Elle a donné lieu à des débats très riches, qui ont abouti à un ensemble de recommandations très cohérentes. L'obligation

dit clairement que, d'un point de vue épidémiologique, la myofasciite à macrophages était une maladie qui n'avait été observée qu'en France, à l'exception de quelques cas. Nous sommes donc en face d'une équipe ayant décrit une maladie qui n'existe qu'en France et n'est pas reconnue par l'OMS et cette équipe sème le doute sur l'imputabilité

L'Organisation mondiale de la santé a produit un rapport sur les adjuvants et a conclu à leur innocuité. Les académies de médecine françaises, le Haut Conseil de la santé publique, toutes les agences de sécurité sanitaire du monde, la FDA américaine, l'Agence européenne des médicaments, qui fonde la pharmacovigilance, concluent à l'innocuité des vaccins à base d'adjuvants aluminiques. Je veux bien qu'en France on continue de douter. Une équipe travaille, ses projets sont financés, elle répond à des appels à projets et personne ne l'empêche de travailler sur ce sujet. Toutefois, à un moment donné, nous devons prendre nos responsabilités. Ces vaccins existent, ils sont efficaces

Cohen ... Il faut financer la recherche publique ! Bien sûr ! Rien n'empêche ces équipes de postuler et d'accéder à des financements de recherche, comme toutes les équipes du monde ! En France, il n'y a pas de recherche avec des financements fléchés.

l'obligation sera effective au 1 janvier 2018, d'autre part, toutes les études de pharmacovigilance. Nous ferons un état des lieux de la littérature, ce qui permettra aux citoyens, aux parties prenantes, aux journalistes, aux élus, de se tenir informés d'un nouvel effet secondaire hypothétique qui surviendrait chez un enfant français. Nous n'empêchons personne de travailler, bien au contraire. À un moment donné, il faut tout de même se rendre

mais d'inciter fortement à la vaccination contre les infections liées aux papillomavirus humains, le HPV, responsable de nombreux cancers génitaux, aussi bien chez les femmes que chez les hommes. est estimé à près de 48 000 par an en Europe. Les auteurs de cet amendement s'appuient sur les recommandations du Haut Conseil pour la santé publique, qui constate une faible couverture vaccinale en France, en dépit d'une efficacité démontrée sur la prévalence des infections à HPV. Le Haut Conseil constate par ailleurs que « les données de pharmacovigilance, internationales et nationales, avec un recul de plus de sept ans, ne permettent pas de retenir l'existence d'un lien de causalité entre cette vaccination et les événements indésirables graves qui lui ont été attribués en France Le Haut Conseil rappelle que la stratégie actuelle de prévention des infections et des maladies liées aux HPV par la vaccination concerne les jeunes filles âgées de 11 ans à 14 ans, les hommes ayant des rapports avec les hommes jusqu'à l'âge de 26 ans, ainsi que les personnes immunodéprimées. Le présent amendement vise donc à augmenter la couverture vaccinale contre le HPV au sein de ces populations, afin notamment d'éviter des cancers

Cette obligation est satisfaite par les dispositions du code de la santé publique relatives à l'information du patient et au consentement éclairé. Elle est également satisfaite par le code de déontologie médicale. La commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, l'avis

33 de l'article 34 est ainsi rédigé : « Une évaluation de l'impact de l'élargissement des obligations vaccinales est réalisée par le Gouvernement chaque année à compter du dernier trimestre 2019. Elle est rendue publique. Or cette disposition a été adoptée par l'Assemblée nationale avec l'exposé des motifs suivant : « Cet à ce que le taux de couverture vaccinale soit évalué chaque année par la Haute Autorité de santé, qui s'appuie sur des données épidémiologiques, des études sur l'efficacité et la tolérance des vaccinations. » Ma question est donc simple : pourquoi ne pas écrire, directement et simplement, que c'est la Haute Autorité de santé qui réalise l'évaluation, puisque telle était bien l'intention initiale du législateur ? J'ajoute qu'au regard de la défiance

de prévention et de promotion de la santé. Santé publique France étant une agence sanitaire placée sous la tutelle du ministère de la santé, le Gouvernement pourrait y recourir pour évaluer chaque année la mise en oeuvre du dispositif prévu à l'article 34. La commission est donc plutôt défavorable à cet amendement, mais Mme la ministre va nous donner son

nous fournir les données de pharmacovigilance. La Haute Autorité de santé, elle, a pour mission d'établir des recommandations vaccinales et de proposer des adaptations du calendrier des vaccinations. Nous avons donc besoin

Les actes obligatoires, en matière de santé, sont en général pris en charge à 100 % ; c'est le cas, par exemple, des visites médicales obligatoires de l'enfant. C'est bien normal : puisque la collectivité pose une obligation, elle doit assurer sa prise en charge.

contre la rougeole, les oreillons et la rubéole, dont la prise en charge à 100 % a été instituée lorsque le ministère et l'assurance maladie, il y a quelques années, ont lancé une campagne pour « booster » cette vaccination, dont le taux de couverture était bien trop bas. Cette prise en charge à 100 % couplée à une campagne d'information- il faut redire l'importance de l'information et de la mobilisation des professionnels de santé -a permis de faire progresser significativement

! Le sujet n'est donc pas là. Et toutes les personnes qui n'auraient pas de mutuelle, aujourd'hui, peuvent aller en PMI ou en centre de vaccination, où ces vaccins seront mis à disposition gratuitement.

y ont eu recours en 2016. Cet amendement vise donc, en cohérence avec les diverses mesures proposées par le Gouvernement pour lutter contre le tabagisme, à autoriser les entreprises qui commercialisent ces traitements à faire la promotion de ce dispositif sous le contrôle de l'ANSM.

La commission comprend tout à fait l'objet de l'amendement : il s'agit de favoriser les traitements nicotiniques de substitution, qui sont assez peu utilisés. Néanmoins, il nous semble que la publicité autour de la prise en charge de ces substituts doit relever de la communication de l'assurance maladie elle-même ou des campagnes de prévention menées par les pouvoirs publics. Il ne nous a pas semblé judicieux que les laboratoires

en tant que ministre de la santé publique, il nous apparaît important que vous puissiez prendre des décisions, organiser des actions, pour éviter que des

et le plan d'actions interministériel amiante, PAIA, dont le suivi est accessible à partir du portail toutsurlenvironnement.fr. Par ailleurs, l'État publie chaque année, en application de l'article L. 221-6 du code de l'environnement et de l'article 26 de la directive européenne du 21 mai 2008, un rapport sur la qualité de l'air, son évolution possible, ses effets sur la santé et l'environnement et les risques qui en résultent. Pour ce qui concerne les pesticides, enfin, plusieurs rapports des corps de contrôle, notamment pour éliminer les substances les plus dangereuses, sont en cours d'élaboration.

à M. Michel Amiel, sur l'article. Nous voici au coeur du futur de notre système de soins. Il s'agit, comme le rappelle la présentation du Gouvernement du 13 octobre dernier, de garantir à tous un accès égal aux soins. Dans la lignée des propositions de ces dernières années, le modèle du médecin unique, disponible en ville comme en zone rurale, s'est totalement érodé. Les nouvelles organisations doivent répondre au défi que pose la démographie médicale, mais aussi améliorer la prise en charge des patients dans un parcours de soins cohérent. Je dis bien « cohérent » : c'est là l'une des clés pour diminuer les actes redondants ou inutiles- un rapport de l'OCDE montrait que de tels actes représentaient 30 % du total, ce qui est tout à fait considérable. Les équipes pluriprofessionnelles constituent bien une piste qu'il convient de développer, mais il faudra aller encore plus loin. Cette orientation doit également accompagner une transformation profonde de la vision de notre système de santé, jusqu'à présent un peu trop hospitalo-centrée.

C'est essentiel pour mieux appréhender la séquence des soins. Toutes ces organisations nouvelles, j'en suis sûr, ne pourront se construire sans l'association des élus locaux, qui connaissent le mieux la réalité de leur terrain.

pour développer des expérimentations innovantes. Comme vous le savez, mes chers collègues, la loi de modernisation de notre système de santé a décidé de la mise en place de nouveaux PRS,

nous vous avons alertée, en juin dernier, par un courrier resté hélas sans réponse, sur l'élaboration de ces « Nous avions relevé, dans nos départements respectifs, Pas-de-Calais et Val-de-Marne, que ces PRS étaient en train de s'élaborer dans la plus grande discrétion, pour ne pas dire opacité, loin des objectifs de démocratie sanitaire. Pour l'Île-de-France, que je connais mieux, le calendrier officiel indique que les parties prenantes, instance de démocratie sanitaire, collectivités, professionnels de santé, citoyens, doivent être associées à ce processus d'élaboration entre janvier 2017 et mars 2018. Malheureusement, je peux attester que personne, ou presque, n'est au courant de cette démarche. Des Des directeurs d'hôpitaux interrogés avouent, embarrassés, être informés, au mieux, des orientations prises, mais en aucun cas associés dans une démarche de coélaboration. Les enjeux sont pourtant fondamentaux, et il me semble regrettable que l'on se prive de compétences variées et complémentaires, existant sur les territoires, privilégier une vision purement technocratique. Certes, un projet de cadre d'orientation stratégique élaboré par l'ARS a été soumis à la conférence régionale de la santé et de l'autonomie. Ces deux instances sont évidemment légitimes, mais il faut reconnaître que leur composition et leur fonctionnement ne sont pas des plus démocratiques ni des plus représentatifs. Aussi avons-nous le sentiment que ce projet de cadre d'orientation stratégique a été élaboré de façon restreinte, et que les choses échappent au plus grand nombre, y compris aux parlementaires que nous sommes. quant à elles débuter courant janvier 2018 ; mais là encore, j'ai quelques craintes. Pouvez-vous nous rassurer, madame la ministre, sur ces différents points, et nous dire que les PRS2 ne seront pas élaborés sans faire vivre de façon élargie la démocratie sanitaire ? La parole L'article 35 prévoit un cadre d'expérimentation pour l'innovation dans le système de santé, visant à favoriser l'émergence d'organisations innovantes dans les secteurs sanitaire et médico-social, ou à améliorer la pertinence des prescriptions médicamenteuses. Il précise les modalités de pilotage et de financement d'un tel cadre. Pour notre part, nous avons des propositions alternatives pour l'innovation dans le système de santé : une vision large, prospective et partagée à repenser le système de santé et l'hôpital public, afin de répondre aux besoins de santé d'aujourd'hui et de demain. Comment, en effet, affronter le développement intolérable des inégalités sociales, le vieillissement de la population, le développement des maladies chroniques, celui des technologies biomédicales ou du numérique ? Selon nous, il faut partir des besoins de proximité, des exigences de qualité et de sécurité, organiser les coopérations, afin de

de construire de véritables coopérations pour assurer la continuité des soins, replacer l'hôpital de proximité dans un maillage de services de santé publique de proximité, avec un réseau de centres de santé public et non lucratif. En somme, il s'agit de construire une politique publique et territoriale de santé. Aussi l'organisation des soins sur un territoire devrait-elle se faire en associant la population à la définition des besoins locaux. Dans ce dispositif, la place des centres de santé doit être revalorisée ; ils doivent être développés et encouragés. Ce sont des structures de soins ambulatoires de premier recours et de second recours. Ils peuvent être médicaux, dentaires, infirmiers ou polyvalents ; ils sont créés et gérés par des organismes à but non lucratif, des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale ou des établissements de santé. Ils ne pourraient, à l'avenir, être adossés à des sociétés commerciales à but lucratif- l'une

un cadre d'expérimentation pour l'innovation dans le système de santé. Nous espérons son succès, pour la France et nos territoires, pour les déserts médicaux, les hôpitaux ou les cliniques. Renforcer l'offre de soins est toute l'ambition de l'article. Notre groupe souhaite apporter tout son soutien aux mesures de meilleure coordination du parcours de santé, d'amélioration de la prise en charge sanitaire et médico-sociale ou de développement des modes d'exercice regroupé. Je pense d'abord au renforcement matériel de l'offre de soins, avec une meilleure identification des zones déficitaires,

qui ouvre la voie à l'expérimentation en matière d'organisation de soins, de lien entre établissement et ville, de nouveau mode de rémunération et de partage de tâches. Sur ce dernier point, les infirmières- j'ai l'habitude de parler au féminin -sont les premières concernées, avec ce que l'on appelle les délégations de tâches.

Craignant que l'exécutif actuel, malgré des déclarations d'abord volontaristes, ne fasse de même, nous avions décidé de replacer cette question d'égalité, mais aussi de santé publique, au coeur du débat politique. cela que vous en parlez ! ... en application du fameux article 40 de la Constitution, au motif qu'il prévoyait la prise en charge par l'assurance maladie de l'assistance médicale à la procréation ouverte aux couples de femmes, créant ainsi une charge publique. Cette décision appelle, me semble-t-il, plusieurs commentaires. Si l'on considère l'ouverture de la PMA à toutes les femmes comme un enjeu d'égalité, il convient évidemment que celle-ci soit prise en charge par l'assurance maladie, comme elle l'est pour les couples hétérosexuels. Nous avions donc pris soin de gager la dépense en prévoyant une hausse de la taxation du tabac, responsable, au même titre que les pesticides, le bisphénol A, les perturbateurs endocriniens et le stress, de la baisse de la fertilité. Pour cet amendement, le gage n'a pas suffi, et le président de la commission des finances, sans motiver plus avant sa décision, a purement et simplement supprimé cette question des débats. Or l'interdiction de l'accès à la PMA, si elle relève au mieux de l'hypocrisie, au pire de la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle, a également d'importantes répercussions sur le plan sanitaire.

le 6 novembre dernier sur un site internet. Elle a été élaborée avec l'ensemble des parties prenantes. Les ARS pourront travailler sur leurs projets régionaux de santé

s'élaborent avec les parties prenantes, les fédérations, les professionnels de santé, mais également les conférences régionales de santé et d'autonomie, donc avec l'ensemble des associations.

dans le plan d'accès territorial aux soins, j'ai indiqué que nous doublerions le nombre de maisons de santé pluriprofessionnelles et/ou de centres de santé. Après tout, que l'exercice soit salarié dans un centre de santé ou

restreint. Somme toute, c'est plutôt rassurant, puisqu'ils doivent offrir le tiers payant obligatoire pour tout le monde, être à tarifs opposables, c'est-à-dire sans dépassement d'honoraires, et avoir une gestion désintéressée, c'est-à-dire un réinvestissement des bénéfices. des bénéfices. Je souhaite enfin répondre à M. Daudigny sur les délégations de tâches. Vous le savez, les « protocoles 51 » tels qu'ils avaient été prévus par la loi HPST ne fonctionnent pas. Ils sont très longs à mettre en oeuvre. La Haute Autorité de santé est très peu saisie sur le sujet et met du temps à répondre. Ces protocoles ne se déploient pas. C'est la raison pour laquelle je souhaite que le plan d'accès territorial aux soins permette des délégations de tâches sur les territoires sous-dotés. Cela se fait déjà. Or ces infirmières ne sont pas couvertes. Pourtant, elles adaptent des INR, des traitements. Il faut donc les couvrir avec des protocoles qui seront validés dans le cadre des expérimentations. Par

En effet, les expérimentations autorisées par l'article 35 devraient précisément permettre d'aboutir à la structuration de parcours de santé assurant une meilleure articulation entre les différents intervenants, qu'ils exercent en ville, en hôpital ou dans le secteur médico-social. Il ne nous a donc pas paru utile de figer une définition dans la loi ou de prévoir des expérimentations « génériques » sur la notion de parcours de santé. Cela semble redondant avec les objectifs déjà fixés dans le texte.

Cela nécessite aussi une nouvelle organisation et des innovations dans le système de soins. Ainsi, sur la question de la délégation de tâches, qui vient d'être abordée, les consultations-conseils doivent se développer et de nouveaux outils doivent être mis en place. Je propose donc

comprend en effet l'importance de ces sujets. Toutefois, il nous a semblé qu'un tel ajout conduirait à élargir le champ des expérimentations à l'ensemble de la politique de santé. Il paraît préférable, pour ne pas trop se disperser, de s'en tenir aux objectifs, qui sont déjà ambitieux coordination des parcours et amélioration des prises en charge et de l'accès aux soins. Le cadre expérimental ne fera pas obstacle à la possibilité pour les ARS de continuer à financer des actions en la matière dans le cadre du fonds

organisationnelles et d'impulser une réflexion sur leur possible généralisation.

Il est ainsi proposé que les centres départementaux de l'enfance, les CDE, et les maisons d'enfants à caractère social, les MECS, puissent créer des unités d'une dizaine de lits permettant de prendre en charge rapidement des mineurs souffrant de troubles du comportement.

d'enfants à caractère social au-delà de 18 ans. Il s'agit d'assurer une transition en douceur du suivi de ces jeunes au-delà de la majorité. Les départements ne peuvent malheureusement plus financer de telles démarches. Ils se désengagent des contrats jeunes majeurs,

après l'alinéa 8. Je vous propose de prendre en compte l'amélioration des conditions de travail des professionnels de santé, quel que soit leur statut, et des professionnels du champ médico-social.

sommes tous particulièrement conscients de l'importance du phénomène de, notamment chez un certain nombre de professionnels qui exercent dans des conditions difficiles. Dans notre volonté commune de mettre en place un système de soins fonctionnant de manière plus satisfaisante, la prise en compte de l'amélioration des conditions de travail des professionnels de santé me semble devoir être considérée comme prioritaire. Quel

coconstructeur de l'évolution du système de santé.

but de décliner toutes les maladies les unes après les autres. En revanche, j'ai donné des instructions très claires à l'assurance maladie, dans le cadre de la convention qui est en train d'être renégociée avec les dentistes,

Comme le recommande la Cour des comptes depuis 2015, un forfait unique, adapté au profil de chaque patient remplaçant les seize forfaits de rémunération en vigueur, permettrait de réformer le financement de la dialyse, et par là même de développer la dialyse à domicile, solution préconisée par les différentes agences de santé et demandée par beaucoup de patients. Ce forfait comporterait des majorations et des minorations en fonction notamment du profil du patient et des résultats des traitements. Les frais de transport, examens biologiques, supplémentation nutritionnelle destinée à remédier aux carences liées au traitement et une part de paiement à la performance y seraient intégrés. Cela reviendrait à créer, tout d'abord, un forfait de suivi hebdomadaire pour les néphrologues, qui sera le même, quelle que soit la technique de dialyse utilisée ; et ensuite un forfait hebdomadaire de traitement de l'IRCT, l'insuffisance rénale chronique terminale, par dialyse pour les établissements, indépendamment de la thérapie, le tarif étant basé sur la charge en soi dont a besoin chaque patient. Nous sommes face à une demande des patients. La réforme de cette tarification marquerait une étape importante. Quel

de remédier à cette difficulté. Ce qui est important chez l'optométriste, c'est qu'il a suivi cinq années d'études après le baccalauréat et qu'il a toutes les compétences nécessaires pour mesurer les corrections à apporter à un défaut de vision.

à travailler avec les différentes filières. Il s'agit plutôt de protocoles de coopération entre professionnels. Or l'article 37 du PLFSS vise à accélérer l'examen des déploiements des protocoles de coopération qui relèveront des priorités ministérielles.

Les modifications apportées aux règles de rémunération dans le cadre des expérimentations auront pour objet de promouvoir un recours plus pertinent aux produits de santé.

mentionnés à l'article L. 165-1 et la qualité des prescriptions, en modifiant : a) Les conditions de prise en charge des médicaments [ ...] ; b) Les modalités de rémunération ». L'article 35 a donc pour but de mettre en place des incitations financières

d'une modulation en lien avec la prescription ou l'usage d'un médicament. L'objectif est d'être incitatif et de renforcer le bon usage ou la limitation de la prescription.

de financement de la sécurité sociale pour 2018 visent à développer une meilleure prise en charge du patient. Il est toutefois important d'adosser ces expérimentations à un établissement de santé ou à une structure ayant la personnalité morale pour ainsi ancrer juridiquement l'expérimentation, par exemple

L'introduction de cette mesure risque de créer un précédent dangereux en matière de santé publique, en permettant à des personnes non professionnelles de santé de dispenser un médicament au domicile des patients. Or, si tant les prestataires que les pharmaciens peuvent être compétents pour installer le matériel nécessaire à la dialyse, seul le pharmacien a la responsabilité pleine et entière de la dispensation de médicaments. Ce dernier est donc seul compétent pour dispenser le dialysat au domicile des patients.

la loi HPST et introduit par un décret d'avril 2011 dans le code de la santé publique. Ce statut permet aux officinaux d'intégrer les différentes organisations pluriprofessionnelles renforçant la coordination des soins. soins. Pour permettre un réel développement du pharmacien correspondant, il est important de faciliter la mise en oeuvre pratique des protocoles de soins. Cela rejoint la priorité n° 3 de votre engagement, madame la ministre, qui est de renforcer l'accès territorial aux soins, c'est-à-dire de favoriser une meilleure organisation des professions de santé. Cela permettra également de libérer du temps médical. En effet, il s'agit bien ici de coopération entre le pharmacien correspondant et le médecin traitant. C'est donc à la demande du médecin, ou avec son accord, que l'on pourra adapter un traitement chronique. L'amendement

L. 4211-1 du code de la santé publique sur le monopole des pharmaciens. Une telle dérogation était déjà prévue par l'article 43 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014, autorisant des expérimentations en vue d'améliorer le parcours de soins et la prise en charge des personnes atteintes d'insuffisance rénale chronique. Elle vise à permettre l'intervention de prestataires pour assurer des dialyses à domicile, susceptibles d'améliorer la prise en charge des patients et leur qualité de vie. Il est explicitement prévu que cela doit se faire sous la responsabilité d'un pharmacien, ce qui constitue une garantie nécessaire.

pour valoriser, certes légitimement, la fonction de pharmacien correspondant. Quant à l'amendement n° 220, il pose la question des conflits d'intérêts et vise à encadrer l'intervention à domicile des prestataires pour la pratique de dialyses. Le cahier des charges des expérimentations apporte probablement des réponses à ce sujet. Si nous partageons son objectif, nous voyons que la dérogation prévue dans le texte suscite en pratique de nombreuses questions, sur lesquelles la commission a souhaité avoir des assurances. Nous demandons donc l'avis du Gouvernement sur ces trois amendements.

pour 2014. Elle permet aux prestataires d'intervenir à domicile pour dispenser les dialysats et autorise ainsi une prise en charge à domicile des patients. Les prestataires ne sont normalement pas autorisés à dispenser de tels produits. C'est pourquoi cette dispensation est effectuée sous la responsabilité d'un pharmacien.

387 rectifié . Une réflexion sur l'évolution des compétences des pharmaciens d'officine est d'ores et déjà engagée avec l'assurance maladie dans le cadre conventionnel, conformément aux dispositions prises

dans le système de santé prévues à l'article 35 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018. Il peut s'avérer indispensable de déroger aux règles qui déterminent les champs de compétence des professionnels de santé. Il est proposé

Les protocoles de coopération introduits par l'article 51 de la loi HPST permettent déjà de déroger à la répartition des compétences entre professionnels de santé. santé. Même si le cadre juridique de ces coopérations est lourd, comme l'a souligné en 2014 un rapport rédigé par Alain Milon et Catherine Génisson, il a au moins le mérite d'exister. En outre, l'article 37 du projet de loi ouvre des possibilités de tarification d'actes en équipe et accélère

Le présent amendement vise donc à étendre la composition du comité technique aux représentants des professionnels de santé, acteurs incontournables du système de santé et dont les opinions doivent être prises en compte.

ayant pour but d'assurer un suivi des expérimentations. Ce comité n'intègre cependant aucun représentant de l'hospitalisation privée. Il est donc proposé de définir sa composition par décret et d'y associer les fédérations hospitalières, publiques comme privées, qui sont pleinement qualifiées pour apporter leur expertise de terrain sur les projets d'expérimentation.

La finalité des expérimentations et de leur évaluation doit bien être leur éventuelle généralisation, par leur transcription dans le droit commun.